modifié, l'ensemble de la proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d'organisation de l'élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19. Il a été décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune. Mes chers collègues, notre séance se tient aujourd'hui salle Médicis, selon les mêmes règles que dans l'hémicycle. Aussi, je vous invite, pour la discussion des articles, à vous lever et à utiliser les micros installés au bord des travées pour vos prises de parole. Dans la discussion générale commune, la parole est à M. Philippe Bonnecarrère, auteur de la proposition de loi organique et de la proposition de loi ordinaire. Madame la Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la vie démocratique continue et nous siégeons ce matin dans

apanage des régimes démocratiques, alors que la guerre est là, en Europe, que des hommes meurent sous les tirs de missiles ou les obus d'artillerie. Tout reste à faire afin que l'Ukraine ne soit pas l'équivalent des Sudètes pour l'Europe de 2022. Les dispositions proposées ne portent aucune modification substantielle de nos règles électorales, de type parrainages ou vote par correspondance ou électronique. Elles visent simplement à adapter certaines règles de droit électoral au contexte sanitaire lié à l'épidémie du covid-19 : possibilité de se voir confier des procurations, modalités plus aisées d'établissement des procurations à domicile, possibilité accordée aux préfets de dédoubler les bureaux de vote si les communes le souhaitent, enfin, ce qui est peut-être le plus important d'un point de vue pratique, renforcement de la couverture de la campagne électorale

les mesures qui vous sont proposées, vous les connaissez. Elles ont été utilisées pour l'essentiel lors des élections municipales de 2020 et des élections départementales et régionales de 2021. Le Gouvernement n'a rien prévu au mois de décembre 2021, lorsqu'il a préparé ses mesures sanitaires. Nous n'avons pas eu le droit d'amender le texte, puisqu'il s'agissait d'une matière organique, et le Gouvernement n'a pas plus souhaité le succès des propositions que je vous présente en refusant, alors que cela lui a été expressément demandé, d'accélérer leur examen.

texte comporte simplement l'intégration de dispositions légales qui avaient été adoptées durant le quinquennat. Pour lever le moindre doute, je renvoie aux déclarations de Mme la ministre ici même, au Sénat : « Le projet de loi organique que vous examinez ce soir nous invite, pour sa part, à renouer avec une forme de " normalité démocratique tout en nous projetant résolument dans l'avenir. » Elle évoquait également un peu plus loin la nécessité de se « projeter collectivement au-delà de la crise sanitaire- dont nous espérons tous que, grâce au vaccin, elle sera derrière nous en 2022

Cette règle ne s'est jamais appliquée aux opérations techniques de campagne ou de vote. Mes chers collègues, si vous avez le plus petit doute, reportez-vous aux élections municipales : nous avons adopté le dédoublement des procurations par la loi du 22 juin 2020

Le texte que nous soumettons à votre examen a finalement la nature d'un appel, un appel au pluralisme et un appel très modeste, j'en conviens, par les propositions techniques avancées, en faveur d'une lecture plus équilibrée de nos institutions.

malgré la conjoncture internationale. Nous examinons la proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d'organisation de l'élection ainsi que la proposition de loi visant à améliorer les conditions sanitaires d'organisation des élections législatives dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19, présentées par notre collègue

Ces deux textes proposent des éléments de réponse à des questions que le pouvoir exécutif a apparemment choisi, de manière assez difficilement compréhensible, de ne pas aborder. Le Gouvernement n'a en effet prévu aucune mesure pour tenir compte du contexte sanitaire adapter les modalités d'organisation des scrutins à venir, pourtant majeurs pour la vie démocratique de notre pays. Cette absence d'anticipation semble d'autant moins compréhensible que le Gouvernement,

La persistance de l'épidémie de covid-19 pourrait en effet faire peser un risque important aussi bien sur la participation des électeurs aux scrutins présidentiel et législatifs que sur la sécurité sanitaire des personnes chargées de les organiser. Par ailleurs, la question des conséquences de l'épidémie sur le déroulement de la campagne électorale et sur la tenue des meetings politiques et, plus généralement, la question de la couverture audiovisuelle de la campagne méritent également d'être posées.

Il en va ainsi de l'assouplissement des conditions de vote par procuration, qui passe par deux dispositions : l'ouverture du droit à la double procuration, d'une part, la facilitation de l'établissement des procurations à domicile, d'autre part.

Cette mesure revêt un intérêt pratique indiscutable en facilitant, pour les électeurs ne souhaitant ou ne pouvant pas se déplacer au bureau de vote le jour de l'élection, la recherche de mandataires. Très concrètement, elle permet par exemple à un électeur de disposer d'une procuration pour ses deux parents ou ses deux grands-parents. De manière quelque peu surprenante, si personne, je crois, parmi les élus et électeurs, ne conteste la pertinence d'une telle mesure, l'obstacle qu'oppose le ministère de l'intérieur est d'ordre technique Le répertoire électoral unique, opérationnel, je le rappelle, depuis le 1 janvier 2022, a été en effet paramétré pour n'accepter qu'une seule procuration établie en France- un choix curieusement déconnecté de toute considération sanitaire et pratique, puisque nous sommes en pleine pandémie En tout état de cause, il ne revient pas au Parlement de légiférer en fonction des difficultés techniques qui se poseraient au ministère de l'intérieur en raison de son propre manque d'anticipation. C'est pourquoi la commission a adopté cette disposition de bon sens. liées à l'établissement des procurations à domicile sont aujourd'hui strictement encadrées. L'électeur doit en effet accompagner sa demande d'une attestation sur l'honneur de son incapacité à se déplacer dans une brigade de gendarmerie en raison d'une maladie ou d'une infirmité grave ; il ne peut exprimer sa demande que par écrit. Les propositions de loi organique et ordinaire visent à reprendre le même dispositif que celui qui a été prévu lors du second tour des élections municipales de 2020, afin d'apporter à l'électeur plus de souplesse et de simplicité que ne lui offre le droit existant. Ainsi, toutes les personnes vulnérables qui souhaitent éviter de prendre le risque d'une contamination pourront établir ou retirer une procuration depuis leur domicile. La commission a également adopté cette disposition, qui permettra elle aussi d'éviter que le contexte sanitaire ne constitue un frein à la participation électorale. Par ailleurs, afin d'éviter une trop forte concentration des électeurs dans les bureaux de vote, les propositions de loi visent à ouvrir aux préfets la possibilité d'augmenter le nombre de bureaux de vote. Il s'agit là d'une mesure proposée par la commission des lois au mois d'octobre 2020

Aujourd'hui, le code électoral oblige les préfets à fixer le périmètre des bureaux de vote avant le 31 août de l'année précédant le scrutin. Avec la disposition prévue par les deux propositions de loi, ils auront la possibilité, après cette date, de dédoubler ces bureaux de vote dans les communes. Il s'agit là d'un outil supplémentaire.

C'est d'autant plus important que nous nous trouvons à six semaines d'une élection extrêmement importante pour la vie démocratique de notre pays et que tous les candidats ne sont pas officiellement déclarés. À cette fin, la commission a préféré substituer l'obligation, pour l'ensemble des candidats, de débattre entre eux avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il appartiendra bien sûr aux candidats et aux différentes chaînes de s'entendre sur les modalités concrètes d'organisation et de

Vous le savez, ce n'est pas une surprise : l'avis du Gouvernement est défavorable. L'intention du groupe Union Centriste est de favoriser une plus forte participation électorale ainsi qu'une campagne de qualité

on ne revient pas sur le cadre juridique d'une élection à une échéance trop rapprochée de celle-ci, sauf s'il existe des conditions d'urgence absolument exceptionnelle pour prendre de telles mesures. Nous ne souhaitons pas déroger à ce principe. La situation sanitaire de ce mois de février 2022 diffère- et c'est heureux -de ce que nous avons pu connaître lors des élections municipales, communautaires, départementales et régionales de ces deux dernières années. En effet, le contexte sanitaire évolue positivement. Grâce à la responsabilité collective des Français, grâce à notre fort taux de vaccination, nous pouvons désormais appréhender sereinement la tenue des élections sans que paraissent nécessaires des mesures électorales particulières. La poursuite des opérations de vaccination l'application des protocoles sanitaires appropriés garantiront un déroulement régulier de la campagne électorale et des opérations de vote en tant que telles. Je tiens également à vous rappeler que le Premier ministre a mis en place un comité de liaison animé par Jean-Denis Combrexelle, qui réunit régulièrement les administrations impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle ainsi que les candidats et les chefs des formations politiques. Ce comité de liaison doit nous permettre de faire face aux éventuelles évolutions sanitaires, en y apportant des réponses adaptées. Le travail de ce comité a ainsi abouti à l'élaboration d'un protocole sanitaire consacré aux réunions et meetings politiques, partagé par l'ensemble des candidats et partis. Dans ce contexte d'amélioration de la situation sanitaire, la possibilité pour un mandataire d'être détenteur de deux procurations ne nous apparaît pas comme une mesure nécessaire.

La procuration demeure néanmoins un outil important de facilitation du vote pour ceux de nos concitoyens qui ne pourront pas se rendre physiquement au bureau de vote les jours du scrutin. Je souhaite souligner les efforts engagés par le Gouvernement pour simplifier cette procédure. Le portail www.maprocuration.fr permet, depuis 2021, de rédiger très rapidement sa demande de procuration en ligne. Surtout, depuis le 1 janvier 2022, il est également possible, grâce au répertoire électoral unique, de donner procuration à un électeur qui n'est pas domicilié dans la même commune. C'est une avancée majeure, qui apportera une plus grande souplesse dans l'établissement des procurations et dans la recherche d'un mandataire. Enfin, chacun peut demander, sans justificatif médical, la venue à son domicile d'une personne habilitée à établir la procuration. Ces avancées seront pleinement applicables pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Elles répondent à mon sens aux préoccupations exprimées par ces deux propositions de loi. Pour les citoyens qui, dans ce contexte sanitaire, rassurés, des aménagements existent et sont effectifs. En ce qui concerne la possibilité de modifier le périmètre des bureaux de vote, il convient de rappeler que les limites des bureaux de vote sont arrêtées par le représentant de l'État, sur proposition du maire, au 31 août de chaque année pour l'année suivante en application de l'article R. 40 du code électoral. Depuis le début de la pandémie, les préfets et les maires ont été sensibilisés à la nécessité de choisir des lieux de vote permettant de garantir la sécurité sanitaire des membres des bureaux de vote et des électeurs. Cela a permis la bonne organisation des élections départementales et régionales en 2021, alors même que la concomitance de ces deux scrutins conduisait à dédoubler le nombre de bureaux de vote. La tenue des bureaux de vote sera, comme pour les précédents scrutins, soumise à un protocole sanitaire communiqué aux maires. Les bureaux seront par ailleurs dotés en équipements sanitaires. J'ajoute que changer les bureaux de vote à ce stade de l'année, alors que les cartes électorales ont été envoyées, pourrait entraîner beaucoup de confusion

Enfin, j'en viens à la proposition d'imposer l'organisation d'un débat entre l'ensemble des candidats avant le premier tour du scrutin présidentiel. Nous considérons que toute modification du cadre juridique des services de radio et de télévision en période électorale

Je réaffirme ici la détermination du Gouvernement à permettre l'organisation des élections présidentielle et législatives dans les meilleures conditions possible. Le débat que nous avons aujourd'hui porte sur des enjeux importants et je crois que les sujets évoqués pourront nourrir la réflexion pour les prochains scrutins.

pour leur rappeler les modalités pratiques du vote et son importance pour décider de l'avenir de notre pays. Le vote est un droit civique ; c'est aussi un devoir citoyen.

Alors que la crise internationale et européenne dans laquelle nous sommes entrés après l'agression de l'Ukraine n'incite pas aux grands effets de tribune, il est utile de commencer par rappeler que la démocratie joyau, que la paix est un bien commun précieux et que les peuples ont soif de participer au plus près à la vie collective apaisée de leur pays. Les problématiques d'organisation liées à la pandémie et la baisse constante de participation aux élections, y compris municipales, avaient amené à prendre des mesures modificatives des conditions de vote pour les récentes élections départementales et régionales. Ce texte s'en inspire. Les taux d'abstention de plus en plus importants traduisent une remise en question de l'utilité du vote. Nous devons les étudier finement. Le taux d'abstention de la tranche des 18-30 ans figure parmi les plus élevés, ce qui conduit à leur sous-représentation dans les préférences collectives exprimées. De 25 à 44 ans, un peu plus de 90 % des personnes ayant un diplôme de niveau supérieur au bac sont inscrites sur les listes électorales, soit 30 points de plus que les personnes sans diplôme. Ces inégalités devant le scrutin conduisent à des phénomènes de « mal-représentation ». Le manque de confiance envers la classe politique est malheureusement établi, mais cela ne veut pas dire pour autant que les Françaises et les Français ne s'intéressent plus à la vie publique. Pétitions, grèves, manifestations, militantisme de terrain montrent qu'il y a implication et que l'on ne peut pas uniquement parler de repli sur la sphère privée ou d'apathie politique. Notre système électoral est à repenser, pas simplement pour les prochaines échéances ou en raison d'une crise sanitaire. C'est nécessaire, même si ce ne sera pas suffisant. Abaisser le droit de vote à 16 ans doit faire partie de nos réflexions. La jeunesse s'exprime déjà dans les marches, dans les rassemblements. Le droit de vote permettrait à plus de jeunes de s'engager dans la vie politique, alors qu'ils sont les plus concernés par les décisions ou les non-décisions prises sur l'environnement ou la dette. En cette En cette période particulièrement difficile pour les jeunes du fait de la crise du covid, qui a conduit à une précarisation extrême et accélérée de certains, leur participation démocratique à la vie politique semble essentielle et doit être encouragée. J'ai pu noter que cet hémicycle appréciait le fait que les adolescents de plus de 16 ans soient responsables pénalement de leurs actes. Ils peuvent aussi tenir un fusil pour chasser. Ils devraient également être en droit de tenir un bulletin de vote. Notre groupe s'inquiète comme vous de la désaffection électorale, phénomène constant depuis plusieurs années, mais qui a été exacerbé par le comportement de ce gouvernement face aux demandes de plus de démocratie des Français, face aux espoirs suscités par les annonces d'un Président de la République qui se trouve en difficulté

Nous avons un besoin de changement réel : comptabilisation du vote blanc, part de proportionnelle pour les élections législatives- encore une promesse non tenue du candidat Macron de 2017 ... J'insisterai enfin sur le retour à une décorrélation des élections présidentielle et législatives, ces dernières étant devenues un simple vote de confirmation. Cette volonté d'asservir le pouvoir législatif à l'exécutif relève d'une idéologie de l'exercice du pouvoir très solitaire, où le Parlement dans son entièreté apparaît comme une chambre d'enregistrement des décisions de l'exécutif, comme l'a montré

Sans changement profond de notre système démocratique, de nouvelles crises sociales sont à redouter. La méfiance des citoyens à l'égard de la chose publique ne pourra que s'accentuer. Nous devons prendre en compte à sa juste valeur cette défiance, ce désenchantement.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire pèse depuis maintenant deux ans sur bien des aspects de notre vie quotidienne. Notre travail, nos loisirs, nos relations sociales ont été impactés plus ou moins directement, plus ou moins fortement. Pourtant, nous avons su nous adapter et évoluer au gré des vagues de cette pandémie afin de pouvoir continuer à mener une vie la plus normale possible. Il existe malheureusement une exception : notre vie politique, qui n'a pas su s'adapter, se doter des outils lui permettant de surmonter cette crise.

en cette matière, les élus de terrain que nous sommes savent bien que la crise sanitaire vient s'ajouter à une autre crise, plus profonde et plus ancienne. Notre démocratie est malade et les symptômes sont connus de tous : abstention, perte de confiance dans les institutions et les élus. À titre d'exemple, aujourd'hui, c'est le système de parrainages qui est remis en cause. Au regard de ce constat, pouvons-nous vraiment prendre le risque que la crise sanitaire vienne perturber un grand temps fort de notre V République ? L'élection présidentielle reste à ce jour relativement épargnée par l'abstention, mais qu'en sera-t-il si un pic épidémique se déclenche quelques jours avant le premier tour ? Une faible participation alimenterait à coup sûr les procès en illégitimité et viendrait une nouvelle fois fragiliser un système déjà contesté. À ceux qui voudraient m'opposer la récente décrue j'aimerais leur rappeler que si ce virus nous a appris une chose, c'est que son imprévisibilité force l'humilité. Je m'étonne donc du peu d'initiatives qui ont été prises pour sauvegarder tant la campagne que les opérations électorales. Il s'agit pourtant de mesures de bon sens, qui, de surcroît, ont déjà été appliquées par le passé. Ayons tous en tête le second tour des élections municipales, comme nous y exhorte Philippe Bonnecarrère. Celles-ci ont été précipitamment reportées dans l'impréparation au mois de juin Nous devons en tirer les leçons et adapter notre droit électoral pour pouvoir réagir en conséquence. Tant mieux si la pandémie s'éloigne définitivement, mais il est de notre responsabilité de parer à toute éventualité et, en ce sens, je salue ces propositions de loi de notre collègue du groupe Union Centriste. Je regrette d'ailleurs que le Gouvernement n'ait pas jugé bon d'engager lui-même ces travaux ou, à défaut, la procédure accélérée. Il montre ainsi son souhait d'enterrer nos propositions.

Ainsi, la reconduction de l'assouplissement des règles relatives à la procuration est utile. Il s'agit non seulement de protéger les plus fragiles, alors que l'évolution de l'épidémie dans les mois à venir est incertaine, mais aussi de prévenir les phénomènes d'abstention que la persistance de l'épidémie pourrait favoriser. Je suis d'ailleurs convaincue qu'il s'agit d'un axe sur lequel nous devons progresser. Les Français ne comprennent plus la lourdeur de la procédure qui pèse sur l'établissement d'une procuration quand, dans le même temps, l'immense majorité de leurs interactions avec l'administration peut se faire sur un smartphone depuis leur canapé. Il ne s'agit pas ici de désacraliser le vote, qui doit garder une charge symbolique forte, mais nous devons, sans aucun doute, l'adapter à notre époque, surtout quand on sait que 80 % des 18-25 ans se sont abstenus aux dernières élections régionales. En outre, bien que les réunions politiques ne soient pas soumises aux mesures de jauge ou à la présentation du passe vaccinal, le principe de responsabilité a conduit un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle à limiter leurs rassemblements. Pour autant, l'information des électeurs doit être assurée et chaque candidat doit pouvoir avoir l'opportunité d'exposer ses idées et de convaincre les Français. Il est donc essentiel que ces derniers puissent avoir accès aux programmes et positions défendues par les différents candidats afin d'éclairer utilement leur vote le moment venu. En conséquence, au regard des apports de ces textes à la fois sur la protection de la santé des Français et sur notre vie démocratique, le groupe Union Centriste les votera.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, d'ici quelques minutes, nous allons suspendre nos travaux. C'est donc l'occasion d'une rapide rétrospective. Juin 2020, nous sortons du confinement. La courbe épidémique a chuté et pourrait laisser croire à un virus passager. Nous avions cependant voté un texte pour les scrutins municipaux. Juin 2021, un nouvel espoir, le vaccin est arrivé et devrait vaincre le virus. Nous avions cependant voté un texte pour les scrutins

des dispositions relatives aux procurations, nous n'y voyons pas d'objection particulière, même si nous avons toujours un doute sur la mise en pratique concrète de la mesure visant à autoriser le mandant à confier sa procuration à tout électeur, sans exiger que celui-ci soit inscrit sur la liste électorale de la même commune.

Ce sont eux qui connaissent le mieux les moyens humains et matériels dont dispose leur commune pour mettre en place un tel dispositif. Il ne paraît pas envisageable que les préfets puissent l'imposer, surtout au regard des expériences passées, qui ont largement révélé les difficultés que posait, notamment aux petites municipalités, et encore plus spécifiquement aux villages ruraux, l'augmentation du nombre de bureaux. pas moins que, derrière ces mesures d'apparence technique, nous touchons à des problèmes bien plus profonds. Si nous souhaitons faciliter l'exercice des droits civiques, c'est aussi indirectement dans l'espoir de répondre à une crise aiguë de la citoyenneté dans notre société. La participation aux derniers scrutins locaux était très préoccupante. Ces prochains mois diront si cette tendance au désintérêt de nos concitoyens se confirme. Hélas ! je crains qu'il en soit ainsi, tant que la citoyenneté ne sera pas valorisée dans notre société. pas valorisée dans notre société. Pour le professeur de droit public Bruno Daugeron, il suffit d'observer où sont les files d'attente. Elles ne sont plus dans les bureaux de vote, mais dans des lieux où l'imaginaire social est motivé et suscité, c'est-à-dire dans les centres commerciaux, les cinémas et les événements festifs en tout genre. Si les citoyens ne se saisissent plus du vote comme moyen d'expression d'une opinion, sans doute est-ce aussi parce qu'ils ont perdu l'impression que ce vote pouvait influer sur leur mode de vie.

sur le thème : « Comment redynamiser la culture citoyenne ? » J'espère que la prochaine campagne électorale sera à la hauteur des enjeux, pour ne pas démobiliser encore un peu plus les électeurs. Ces remarques étant faites, et sous réserve que nos amendements soient adoptés, notre groupe

Madame la présidente, madame la ministre,

Alors que le Gouvernement décide de lever une grande partie des restrictions sanitaires d'ici au 15 mars, la situation épidémique n'en demeure pas moins fragile. Un variant ou sous-variant peut surgir et de nouveau tout remettre en question. Nous avons raison de préférer la prudence à la fausse certitude. Nous ne voulons pas reproduire ce qui s'est passé lors des élections régionales et départementales le taux d'abstention a atteint un niveau record de 66,6 % et il est réducteur d'expliquer ces chiffres par le seul désintérêt politique des Français.

de l'article 1 de la proposition de loi organique permettant l'organisation d'au moins un débat entre l'ensemble des candidats avant le premier tour. Certaines personnalités politiques partagent la conviction profonde que leur succès ou leur échec dépend en partie du temps qui leur est accordé dans les médias. Ils n'ont pas tout à fait tort. C'est d'ailleurs pour cela que nous devons veiller à un respect strict des règles régissant le traitement médiatique de la campagne présidentielle. Nous ne pouvons pas ignorer le rôle fondamental des médias audiovisuels

activiste du parti animaliste. Considérée comme une « petite candidate », elle ne bénéficie pas du même traitement médiatique que les autres. Elle mérite pourtant toute sa place dans l'espace audiovisuel. La cause animale devrait faire partie du débat présidentiel. Les médias contribuent à façonner la vie politique de notre pays et concourent grandement au choix final que feront les électeurs. Alors, donnons la possibilité à tous les candidats,

donc la guerre toujours recommencée ! Nous étions beaucoup, je pense, à imaginer que la chute du mur de Berlin ouvrirait une ère

en cette période grave, qui nous place dans une situation terrible.

L'idée qu'il y ait un débat entre les candidats relève du bon sens, bien sûr, mais vous n'ignorez pas qu'il y a un dispositif en cours et que ce dispositif prévoit, chacun le sait, une phase préliminaire, une phase intermédiaire, qui va commencer le 7 mars,

et je vois mal comment on pourrait, en cours de partie, changer la règle du jeu. De toute façon, le texte n'a aucune chance d'être définitivement la question de la double procuration a toujours été pour notre groupe une interrogation. On peut comprendre que cette mesure ait été instaurée pour les élections précédentes,

mettant en cause des fraudes liées au vote par correspondance. Il est vrai que les choses ont évolué depuis lors et que la proposition de loi présentée par Éric Kerrouche

Bref, il y a beaucoup d'idées intéressantes. Vous êtes attaché à ce que la démocratie fonctionne mieux, à ce que notre dispositif électoral soit meilleur,

la réflexion de M. Bonnecarrère et de ses collègues : nous nous abstiendrons donc sur ces textes.

parcourir les écrans pour voir que la campagne électorale est déjà intense dans les différents médias. Et je ne vois pas, pour l'instant, de signes flagrants d'atteinte au pluralisme, dans les conditions que fixe la loi que nous avons revue

ne dispose que d'un certain nombre de bâtiments publics, il n'est pas forcément évident de dégager la capacité d'accueil nécessaire dans de bonnes conditions de sécurité pour le public,

En 2021, les élections départementales et régionales, reportées à cause de la pandémie, ont affiché un taux record d'abstention, de l'ordre de 66 %. Grâce au travail des soignants, au respect des gestes barrières et à une politique volontariste de vaccination, nous commençons à voir le bout du tunnel, et nous espérons tous reprendre une vie normale dans les semaines à venir. Néanmoins, les élections présidentielle et législatives se dérouleront dans une situation toujours impactée par la covid-19. Nous remercions donc notre collègue Philippe Bonnecarrère de nous proposer ces textes, qui avancent des solutions concrètes pour faciliter les conditions d'exercice de la démocratie,

que nous vivons pour les droits de l'homme et les libertés en Europe doit nous rappeler l'importance, pour les enjeux démocratiques, des scrutins présidentiel et législatifs à venir en France.

Philippe Bonnecarrère ont l'avantage de tenir compte des dysfonctionnements et des avancées qui se sont produits lors des derniers scrutins départementaux et régionaux, et d'avancer des solutions

et des bénévoles qui, assesseurs ou présidents, donnent de leur temps pour tenir des bureaux de vote et faire en sorte que ces échéances électorales soient une réussite. Pour cela, il faut que le Gouvernement accompagne les élus locaux dans l'organisation de ces scrutins, notamment par des consignes claires et anticipées. Nous devons, pour ces futurs scrutins, nous inspirer des modalités mises en oeuvre pour les dernières élections locales, qui ont démontré notre capacité à nous adapter à la situation sanitaire, grâce au respect des gestes barrières, à l'organisation matérielle des bureaux de vote ou encore au recours à la double procuration. Nous devons aussi tirer les conséquences des dysfonctionnements, certes récurrents, mais plus nombreux lors des scrutins de 2020, notamment dans la distribution de la propagande électorale. Grandir, c'est apprendre de ses erreurs. Ainsi, dans un premier temps, la double procuration permettrait d'apporter une réponse qui a fait ses preuves. La simplification de la procédure, sa centralisation grâce au répertoire électoral unique et sa dématérialisation sur le site www.maprocuration.fr doivent permettre d'offrir cette possibilité, dans un cadre sécurisé, à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Le recours à un mandataire d'une autre commune est une avancée, qui doit être amplifiée, en période de covid-19, par la double procuration. L'obstacle technique avancé par le Gouvernement démontre le manque d'anticipation des services de l'État et ne peut justifier à lui seul le refus du Gouvernement de maintenir cette possibilité. La technique ne doit pas conditionner la démocratie. Enfin, il n'y a pas de démocratie sans un vote éclairé. L'accès à l'information est essentiel pour aider les électeurs à choisir leur candidat,

source d'information pluraliste. Le terrible échec lors des dernières élections a contribué à affaiblir la participation électorale, déjà largement touchée par une abstention structurelle.

surtout lié aux difficultés d'inscription sur les listes électorales à la suite du déménagement des électeurs. Le changement d'adresse reste un processus complexe, qui oblige à fournir de nombreux justificatifs qui impose une procédure de radiation puis de réinscription, y compris lorsque le changement d'adresse se fait au sein d'une même commune. Aujourd'hui, sept millions d'électeurs sont mal inscrits. La refonte des listes électorales va aboutir à l'envoi de nouvelles cartes d'électeurs, modernisées grâce à un QR code. Mais elles pâtiront des mêmes difficultés d'adressage, ce qui risque d'embouteiller les bureaux de vote

Près de 70 communes en font usage à chaque élection, sans que jamais aucun problème important n'ait été relevé. À l'heure où de nombreuses voix souhaitent le recours

ou encore à Boulogne-Billancourt, le renouvellement ou l'extension du parc de machines à voter est bloqué par une décision qui, je l'espère, fera l'objet d'une révision rapide, afin que nous puissions nous équiper des nouvelles machines à voter électroniques, qui garantissent le secret du scrutin.

en Europe. Le taux d'abstention aux dernières élections régionales, l'année dernière, fut de 66,7 %. C'est un record absolu. Ce chiffre, bien évidemment, interpelle les élus que nous sommes. Élection après élection, la participation diminue, jusqu'à atteindre des niveaux dangereux pour la crédibilité de notre démocratie. Les causes sont multiples et la crise sanitaire n'a rien arrangé. Or, si le vote est un droit- un devoir aussi, pour trop peu d'entre nous -, il nous appartient comme législateurs de tout mettre en oeuvre pour en faciliter l'exercice et inciter nos concitoyens

et 2021. Le premier tour des dernières élections municipales s'est déroulé à la date prévue, le 15 mars 2020, sans adaptation particulière sur le plan sanitaire, en dépit de l'apparition quelques semaines auparavant de la pandémie de covid-19. Le second tour a été reporté au 28 juin et s'est accompagné de mesures éphémères destinées à adapter le droit électoral à la situation sanitaire. le droit à la double procuration a été consacré à titre provisoire par la loi. Le régime d'établissement des procurations à domicile a été considérablement assoupli. Enfin, on a prévu la mise à disposition d'équipements de protection pour les électeurs ainsi que pour les personnes intervenant dans les bureaux de vote. Ces trois mesures ont été reconduites pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021, pour lesquelles, en outre, a été mis à la charge du service public de l'audiovisuel le soin d'assurer la couverture du débat électoral relatif à ces deux scrutins. Il est à noter que deux évolutions importantes du droit des procurations sont entrées en vigueur le 1 janvier dernier, cette fois-ci de manière définitive. D'une part, un électeur peut dorénavant donner procuration à un mandataire inscrit sur la liste électorale d'une autre commune que la sienne. Corrélativement, les procurations sont désormais centralisées dans le répertoire électoral unique, qui contrôle automatiquement l'inscription du mandant et du mandataire sur une liste électorale, ainsi que le plafond de procurations détenues par ce mandataire, afin d'éviter des fraudes. D'autre part, le régime d'établissement des procurations à domicile a été assoupli par un décret du 22 décembre 2021. Si ces deux mesures apportent davantage de souplesse au vote par procuration et peuvent constituer une réponse utile pour les personnes que la situation sanitaire dissuaderait de se déplacer le jour du scrutin, elles ne sont toutefois pas à la hauteur des enjeux sanitaires et démocratiques que soulèvent les élections à venir. Le Gouvernement et sa majorité ont donc adopté une démarche ambivalente au regard de l'adaptation de la législation aux circonstances sanitaires à l'approche des élections. Certaines dispositions législatives ont permis au Gouvernement de prendre des mesures provisoires, mais,, celui-ci a refusé d'ouvrir le sujet électoral au niveau législatif tant lors de l'examen de la loi du 10 novembre 2021 de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Ainsi, alors que le Gouvernement ne paraît pas avoir pris toute la mesure du risque que la persistance de l'épidémie de covid-19 pourrait faire peser aussi bien sur la participation des électeurs aux deux scrutins à venir que sur la sécurité sanitaire des personnes chargées de les organiser, la commission des lois du Sénat a souscrit sans réserve au but poursuivi par ces deux textes. Elle en a adopté les dispositions, ouvrant la possibilité à une même personne de se voir confier deux procurations, assouplissant les modalités d'établissement des procurations à domicile et permettant aux préfets de dédoubler les bureaux de vote en cas de risque épidémique particulier. Elle a aussi mis l'accent sur les obligations qui reposent sur les médias audiovisuels en termes de couverture de la campagne électorale, en imposant la diffusion d'au moins un débat entre l'ensemble des candidats afin de renforcer l'expression du pluralisme. Le contenu de ces propositions de loi reprend d'ailleurs très largement plusieurs mesures proposées par le Sénat dès juin 2020.

réconcilier avec leurs représentants, qui sont la traduction de la démocratie représentative ; les réconcilier avec la parole publique, qui trop souvent se dérobe alors qu'elle engage ; les réconcilier avec leur citoyenneté, qui est l'élément essentiel pour choisir notre destin national.

pour mobiliser les Français qui doivent plus que jamais, compte tenu du contexte international, social, économique et culturel, rester des citoyens faisant nation, et non une somme d'individualités ou de communautés.

le dispositif proposé tendant à permettre au préfet d'augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d'assurer la sécurité sanitaire du scrutin. Nous suggérons que cette décision préfectorale ne puisse être prise qu'à la demande du maire. Vous comprenez bien pourquoi, mes chers collègues : il s'agit de ne pas imposer à des municipalités des conditions matérielles et humaines qu'elles ne pourraient pas assumer. Il faut faire confiance aux élus locaux et leur laisser la possibilité d'initier cette procédure.

voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d'organisation de l'élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19.

Le scrutin est ouvert.

texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi organique visant à garantir la qualité du débat démocratique et à améliorer les conditions sanitaires d'organisation de l'élection présidentielle dans le contexte lié à l'épidémie de covid-19.

le contexte lié à l'épidémie de covid-19. Mes chers collègues, par lettre en date du jeudi 24 février, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mardi 1 mars d'une déclaration, suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution, relative à la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La séance du 1 mars serait en conséquence, en accord avec le Gouvernement, requalifiée comme séance gouvernementale. Ce débat pourrait avoir lieu à partir de Pour ce qui concerne son organisation, nous pourrions prévoir que les orateurs des groupes interviennent selon un ordre suivant l'effectif décroissant des groupes, avec les temps de parole suivants minutes pour le groupe Les Républicains, douze minutes pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, dix minutes pour le groupe Union Centriste, huit minutes pour les autres groupes, trois minutes pour un sénateur non inscrit. La commission des affaires étrangères disposerait d'un temps de dix minutes pour conclure le débat. Le délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat serait fixé au mardi 1 mars à midi. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé.